Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues- je vous prie d'excuser M. le Premier ministre, que je viens d'avoir au téléphone -, nous célébrons cette semaine la francophonie, dont la Journée internationale se tenait hier. C'est la raison de la présence dans notre hémicycle du drapeau de la francophonie et de celui de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À l'invitation de François Paradis, président de l'Assemblée nationale du Québec et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous procédons à cette célébration de concert avec les parlements des pays de la grande famille francophone. Car la francophonie, c'est l'appartenance à une communauté humaine de plus de 200 millions de personnes à travers le monde, c'est un trait d'union entre des cultures et des sociétés très diverses, mais qui ont en partage non seulement une langue, mais aussi les valeurs et les idéaux qu'elle porte : la tolérance, le dialogue, le respect de la diversité et des droits de l'homme. Un mot les résume peut-être tous : la démocratie Je tiens à saluer l'Assemblée parlementaire de la francophonie et tous nos collègues qui y siègent et qui en défendent les valeurs. Je remercie plus particulièrement le vice-président délégué de la section française, notre collègue Philippe Mouiller, Christophe-André Frassa, président de la commission politique, et notre collègue Claudine Lepage, vice-présidente de la commission des affaires parlementaires, pour leur engagement dans ce combat. Mes chers collègues, la langue française est la seconde langue des organisations internationales- il faut parfois combattre pour qu'elle conserve ce rang la troisième langue des affaires, la quatrième langue de l'internet. Ne sous-estimons pas les réalisations et les promesses dont elle est riche. Ne sous-estimons pas l'atout que représente pour nous la francophonie, que nous devons défendre et promouvoir.

L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du Bureau du

Je me félicite que la France, par le biais de votre gouvernement, soit ainsi à la pointe du combat pour la préservation de l'environnement. Malheureusement, le ministère de l'économie et des finances n'a pas été informé à temps de l'initiative. En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, juste avant l'ouverture de la semaine sans pesticide, la majorité parlementaire, avec la bénédiction de Bercy, a adopté un amendement au projet de loi Pacte pour repousser de trois ans, à 2025, l'interdiction de la production en France de pesticides, pourtant interdits d'usage dans l'Union européenne. Vous me rétorquerez que le Sénat avait purement et simplement supprimé cette interdiction, et vous aurez raison. Mais je note que le Gouvernement ne s'était alors pas opposé à ces amendements rétrogrades. Bilan des opérations : la France va continuer à produire pendant six ans des pesticides tellement dangereux pour l'être humain, tellement nocifs pour nos sols, que l'Union européenne les a interdits sur son territoire. La même Union européenne qui tergiverse toujours sur le glyphosate, pourtant reconnu pour la deuxième fois comme cancérigène par la justice américaine. C'est dire le niveau de dangerosité des produits en question. Mais ce qui est dangereux pour les Européens ne l'est visiblement pas pour le reste de l'humanité : la France va pouvoir continuer à empoisonner pendant six ans les agriculteurs des autres continents. Alors que le Président est revenu sur sa promesse de sortie du glyphosate en trois ans, le ministre de l'agriculture confirmait pourtant dans le même temps la dangerosité du produit. Conséquence : la politique du Gouvernement est parfaitement illisible. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin proposer une politique ambitieuse de sortie des pesticides ou bien confier cette mission à la FNSEA et aux industriels phytopharmaceutiques, comme le laisse à penser la signature par le Gouvernement du véritable contrat de dupes qu'est le « contrat de solutions de solutions ». La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le sénateur Gontard, je vous remercie de cette question, qui va me permettre de revenir sur notre ambition en matière de produits phytosanitaires. Cette ambition est forte : nous nous sommes engagés à diminuer l'utilisation de ces produits de 50 % d'ici à 2025, nous avons avancé sur la séparation de la vente et du conseil, qui sera opérationnelle en 2019, et nous avons procédé à l'augmentation de la redevance pour pollutions diffuses, également opérationnelle au 1 janvier 2019. En matière de glyphosate, et vous le savez, la France est le pays qui a poussé l'Union européenne à ne réautoriser cette substance que pour cinq ans et non pour quinze ans, et elle a pris l'engagement de sortir du glyphosate en trois Cet engagement est aussi un engagement d'accompagnement de toutes les filières pour ne laisser aucune d'entre elles sur le bord de la route et pour trouver des solutions permettant une production durable en France sans glyphosate. Ces solutions sont travaillées dans le contrat de solutions avec la FNSEA, mais aussi avec le secteur de la recherche, avec l'APCA, avec tous les acteurs du monde de l'agriculture. En ce qui concerne l'exportation, le récent vote de la loi Pacte à l'Assemblée nationale a décalé à 2025 l'interdiction de production, d'utilisation et de stockage de tous les produits, y compris ceux qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne à avoir pris cette décision d'interdiction. Nous souhaitons que celle-ci soit partagée au niveau européen. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons accepté le décalage jusqu'à 2025, pour pouvoir porter ce sujet à Bruxelles et avoir une politique communautaire offensive en la matière. Nous souhaitons aussi accompagner la filière : au lieu d'aller vers une simple interdiction, nous allons accompagner les producteurs pour qu'eux-mêmes changent leurs pratiques et pour qu'ils puissent proposer aux agriculteurs en dehors de l'Europe des solutions qui n'utilisent plus ces produits. La politique que nous menons est bien une politique ambitieuse de sortie, mais c'est aussi une politique de transformation,

Quelle gloire, monsieur Bocquet ! La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour le groupe socialiste et républicain. socialiste et républicain. Ma question s'adressait aussi à M. le Premier ministre. Depuis le début de la crise sociale, le 17 novembre dernier, vous avez géré dans l'improvisation absolue les réponses au mouvement de contestation ainsi que la sécurisation de ces manifestations. Tout le monde a en tête les déclarations du Président de la République le 10 décembre venant contredire les propos de ses ministres, y compris ceux du Premier ministre, tenus quelques jours auparavant. Le 10 décembre n'a été en fait que le début d'une ère de contradictions et d'improvisation, qui trouve son paroxysme avec l'annonce en conseil des ministres du recours à l'armée pour les manifestations de samedi prochain. Le groupe socialiste avait déposé dès le 3 décembre ses propositions pour sortir de la crise. Cela passait par l'écoute et par un dialogue sincère avec les Français et les élus nationaux et locaux. Nous avions également condamné les violences du 1 décembre, comme les violences dans toutes les manifestations. Mais, enfermés dans vos certitudes, vous n'avez toujours pas trouvé les chemins pour sortir de la crise en quatre mois. En laissant pourrir la situation, en jouant sur l'affaiblissement progressif de la contestation, vous avez offert aux casseurs un terrain propice pour leur violence. Vous êtes les seuls responsables de la situation actuelle. En décidant d'appeler les militaires, vous prenez une très grande responsabilité. C'est vrai ! Vous devez expliquer aux Français dans quel cadre vous comptez les employer, quelles consignes leur ont été données. Seront-ils autorisés à faire usage de leur arme en cas de débordements ? Quelle distinction est faite entre délinquant et ennemi ? Nous avons besoin d'éclaircissements à la suite des déclarations contradictoires de vos ministres. Retirer des militaires de l'opération Sentinelle pour les mettre sur le maintien de l'ordre, c'est aussi affaiblir la sécurité des Français dans les gares, dans les aéroports, sur les marchés face à la menace terroriste. En exposant nos militaires, vous prenez le risque de déstabiliser une institution qui est mobilisée- et y est dédiée -depuis 2015 dans la lutte contre le terrorisme. Voulez-vous réellement prendre le risque d'affaiblir les militaires en les embarquant dans une polémique s'il devait y avoir des blessés par balles, voire pire ?

comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin à la préfecture de police, il n'est bien évidemment pas question que les militaires de Sentinelle soient détournés de leur fonction, qui est de

pas pour avoir tenté de brûler vifs une femme et son bébé ... Non, n'en déplaise aux révolutionnaires de plateaux télé qui, samedi après samedi, proclament avec des trémolos dans la voix que nous vivons dans une dictature, je ne parle pas de la France

Son crime ? Avoir défendu ses clientes, des femmes qui retiraient leur voile en public. Pis, avoir contesté publiquement le port obligatoire du voile

où qu'ils se trouvent, celles et ceux qui, comme elle, mettent en jeu leur propre sécurité pour défendre les libertés fondamentales, pour défendre les valeurs universelles qui fondent notre République, au premier rang desquelles la liberté religieuse, l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la défense. Nasrin Sotoudeh a renoncé à faire appel, car elle croit sa cause perdue mais de très nombreux soutiens, de par le monde, refusent de s'y résoudre, comme en témoignent en France les pétitions qui se multiplient. Monsieur le ministre, ma question est très simple : croyez-vous également sa cause perdue ? cause perdue ? La France va-t-elle intensifier son action afin d'obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Nasrin Sotoudeh ?

telle ; d'une femme condamnée pour avoir défendu les droits des femmes, en particulier celles qui contestent, en Iran, l'obligation de porter le voile islamique ; enfin, parce que Mme Sotoudeh est un symbole. Son engagement lui a valu, en 2012, le prix Sakharov du Parlement européen. Il lui a également valu des arrestations, des peines d'emprisonnement et de multiples pressions. C'est pourquoi, comme vous le savez, le Président de la République a publiquement appelé, à l'occasion de la remise du premier prix Simone-Veil, à la libération C'est pourquoi le Président de la République a souhaité, dans le cadre du G7, la faire, symboliquement, membre du conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

considérables avec l'Iran pour préserver l'accord nucléaire, en dépit du retrait américain. Nous l'avons fait, parce que nous honorons notre signature ; mais l'Iran doit aussi respecter ses engagements, en particulier ceux du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Si nous sommes soucieux de préserver l'accord de Vienne,

Il y a eu une demande de la Cour des comptes ; j'ai moi-même proposé à la commission des finances un rapport relatif au renseignement intérieur et à la préfecture de police. Malgré cela, quatre mois après le saccage de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées sont en ruine. La France veut propager l'image de la paix en Afrique, en Syrie, mais elle est incapable de l'assurer aux Parisiens, à quelques encablures de l'Élysée

à renforcer encore plus cette doctrine. Comme vous le savez- le Premier ministre l'a annoncé -, désormais, tout attroupement qui risque de présenter un caractère violent sera immédiatement dispersé. À l'appui de ces mesures, des arrêtés d'interdiction seront

Monsieur Nunez, le fait que ce soit vous qui me répondiez attire la sympathie de cet hémicycle : nous avons tous compris que vous étiez le prochain fusible ! Ma question s'adressait au ministre de l'intérieur,

Mon propos porte sur la grève des douaniers déclenchée le 4 mars dernier sur fond de Brexit. Ses effets se sont vite fait sentir : des perturbations importantes en gare du Nord sur les Eurostar et un blocage complet de Calais- Calais pris en otage, une fois de plus, une fois de trop ! Ce mouvement de contestation dure depuis près de trois semaines. Des contrôles zélés, sporadiques, effectués au port et au tunnel sous la Manche bloquent de manière insupportable tout déplacement normal sur les principaux axes de circulation. Les conséquences pour le territoire sont désastreuses. Je vous les énumère : des camions bloqués sur les bandes d'arrêt d'urgence, parfois neuf heures des chauffeurs sans information, sans ravitaillement, sans sanitaires ; des résidents qui se voient bloqués à des entrées ou des sorties d'autoroute fermées et non pré-signalées, sans information, sans indication de déviation, sans filtrage. Les salariés accusent des retards sur leur lieu de travail, les artisans ont des difficultés pour atteindre leur chantier, les commerces sont désertés, les sociétés sont en attente de leurs livraisons et les transporteurs locaux sont exsangues et excédés. C'est une perturbation de trop qui sème la colère. Monsieur le ministre, nous l'avons appris au travers de la crise des « gilets jaunes » : laisser pourrir une situation, c'est semer et accentuer le mécontentement. Calais est un point de convergence routier qui fonctionne à flux tendu : on doit le gérer dans son exception. Or l'activité économique du Calaisis et le trafic transmanche sont suspendus au piétinement des négociations entre l'État et ses agents. Nous avons besoin d'un signal fort pouvez-vous présenter les moyens que vous comptez mettre en oeuvre pour arrêter ce mouvement de grève ? La

Nous avons apporté des réponses aux douaniers dans le cadre de la préparation du Brexit, avant ce mouvement, avec la programmation et, dès 2019, la création de plusieurs centaines de postes de douaniers pour faire face au Brexit dans des conditions correctes, sans avoir à retirer retirer des forces douanières en d'autres points du territoire. Depuis le début de ce mouvement, les organisations syndicales représentant les douaniers ont été reçues par le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin et, à plusieurs reprises, par le directeur général des douanes. Nous leur avons proposé deux types de mesure. Une mesure immédiate consiste en une revalorisation salariale de plus de 50 euros nets à compter du 1 juillet prochain pour les 17 000 douaniers, ce qui représente un engagement de 14 millions d'euros. De plus, nous avons proposé aux douaniers d'ouvrir des chantiers complémentaires au sujet des conditions de travail.

Premièrement, les perturbations qui sont le fruit de ce mouvement de grève n'ont absolument rien à voir avec la réalité projetée du fait du Brexit, pour une raison toute simple : les contrôles sporadiques et les mouvements que vous évoquez concernent des sorties du territoire, alors que, dans le cadre du Brexit, nous aurons à contrôler les entrées. Deuxièmement, le Premier ministre a demandé à

le groupe La République En Marche. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Il y a quelques jours à peine, le 8 mars, dans une communion quasiment unanime, nous célébrions la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, nombre d'entre nous ont rendu hommage à ces femmes qui ont mené des combats pour que leurs droits avancent au fil des années. Je pense plus particulièrement à celle qui était à votre place, madame la ministre, Simone Veil. Je pense à elle et au combat courageux qu'elle a mené en 1976, à contre-courant de sa famille politique à l'époque, ... Pas toute ! ... pour que les femmes puissent disposer de leur corps et choisir de donner la vie, ou pas, lorsqu'enfanter n'était pas leur choix. Et la question ? Grâce à Simone Veil, le droit à l'avortement est enfin devenu légal en France. France. Mais ce droit fondamental des femmes de disposer de leur corps est en danger, et pas uniquement aux États-Unis, où des intégristes anti-avortement s'enchaînent aux grilles des cliniques pratiquant cet acte médical. Ce danger est aussi présent ici, en France, et il est de surcroît agité par des médecins. Comment est-il possible que le syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, par la voix de son président, puisse menacer le droit à l'interruption volontaire de grossesse ? Pour faire pression sur vous et sur votre gouvernement, ce syndicat a menacé d'ouvrir une grève des IVG s'il n'obtenait pas satisfaction quant aux dédommagements demandés dans des affaires d'erreurs médicales manifestes. donc de la déontologie médicale pour oser brandir une telle menace ? Le président du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France n'en est malheureusement pas à son premier acte anti-IVG. Il y a quelques mois, en en septembre dernier, il déclarait publiquement qu'il considérait l'avortement comme un crime, se défendant peu après d'afficher là une conviction personnelle.

de nous expliquer quelle est votre position face à de tels agissements, comment vous pouvez nous assurer que vous serez la garante d'un droit fondamental des femmes : le droit à l'IVG, leur permettant de choisir d'avoir ou non un enfant

de loi Santé. Comme vous, nous jugeons ce communiqué du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France totalement scandaleux. Il agite comme menace le refus spécifique d'un acte, et pas n'importe lequel. Le refus de l'interruption volontaire de grossesse est un acte militant, un acte signifiant. Ce n'est pas digne d'un syndicat. Dès que la ministre des solidarités et de la santé a eu connaissance du communiqué dont inadmissible de ces menaces destinées à se faire entendre. Vous l'avez dit, elles vont à l'encontre du respect inconditionnel du droit à l'IVG, garanti dans notre pays. Ces nouvelles déclarations sont inacceptables de la part d'un syndicat qui entend représenter les gynécologues-obstétriciens. Cette profession doit être au plus près des souffrances des femmes et accompagner ces dernières, notamment dans ce moment très difficile et très douloureux qu'est l'interruption volontaire de grossesse. Sachez qu'en aucun cas une telle prise en otage des femmes ne servira de levier de négociation au sein de notre ministère ; en aucun cas une telle prise en otage des femmes ne peut non plus servir à la médiation

territoriales. Dans son rapport annuel publié la semaine dernière, le Défenseur des droits met en garde l'État contre le risque de rupture entre les services publics et les usagers. En 2018, 94 % des réclamations qui lui ont été adressées portaient en effet sur cette relation des usagers avec les services publics. Parmi les premiers sujets de préoccupation figure la dématérialisation des procédures administratives, que le Gouvernement souhaite achever en 2022. D'une part, cette dématérialisation soulève de nombreuses difficultés d'ordre technique et organisationnel : il suffit de se pencher sur la délivrance des titres sécurisés dans les transports pour voir que les exemples de défaillances sont nombreux. D'autre part, comme l'a très justement rappelé mon collègue Jean-Yves Roux au mois de janvier dernier, la dématérialisation des services publics nécessite une large couverture internet, un bon équipement des ménages et une maîtrise de l'outil informatique. Or plusieurs centaines de communes n'ont toujours pas accès à internet et 13 millions de Français sont encore en difficulté avec le numérique, sans compter le coût de l'équipement informatique, que l'on fait bien sûr peser sur les ménages. Le numérique est un facilitateur indéniable dans de nombreux domaines : il n'est pas question de remettre en cause un tel progrès. Mais, dans cette phase de transition, il est essentiel de renforcer l'accompagnement et l'inclusion numérique, car une absence de l'État dans les territoires peut amplifier les difficultés d'accès aux droits et le sentiment d'injustice et d'abandon, notamment en zone rurale, où les services de proximité sont en déshérence. Il existe une fracture territoriale de plus en plus profonde entre la France des métropoles et la France des territoires, qui cumule toutes les difficultés : déserts médicaux, suppression de services dans les hôpitaux et la justice, fermeture d'écoles et de commerces, hausse du coût de la vie, transports en commun inexistants, Ajoutez à cela la disparition des services publics et vous obtenez un terreau fertile pour les extrêmes. Aussi, je souhaite savoir quelles actions le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour reconnecter les territoires et rendre effective la promesse républicaine d'égalité d'accès aux droits. La parole

le sénateur Éric Gold, je partage votre diagnostic : si la dématérialisation de certains services est indispensable pour répondre aux besoins de nos concitoyens, nous devons être très attentifs à la situation des 13 millions de personnes qui ressentent des difficultés dans l'usage du numérique.

aidé en cela par les collectivités territoriales, qui agissent aussi dans les territoires pour développer l'accès au très haut débit d'ici à 2022.

il faut accompagner. À ce titre, la mise en place de mesures fortes d'inclusion numérique, avec le guichet « cohésion numérique des territoires », se traduit par un soutien financier pouvant atteindre 150 euros pour l'installation d'équipements.

ajoute la présence, dans les sous-préfectures et les préfectures, de médiateurs numériques pour aider les usagers. Mais bien sûr ... Monsieur le sénateur,

Ma question s'adressait initialement à M. le Premier ministre. Depuis quelques jours, nous assistons à une véritable cacophonie de la part de ce gouvernement, sur fond de réforme des retraites. Alors que la concertation préalable à cette réforme touche à sa fin, alors que depuis le début il a toujours été établi que le recul de l'âge de la retraite n'était pas à l'ordre du jour, voilà que les ministres jouent des partitions différentes. Mme la ministre des solidarités et de la santé en affirmant que le sujet n'est pas tabou. S'ensuit, de manière fort légitime, l'étonnement du Haut-Commissaire, pour qui cette question ne faisait pas partie du cahier des charges, si j'ose m'exprimer ainsi. Après un rétropédalage de Mme la ministre des solidarités et de la santé, c'est au tour du porte-parole du Gouvernement d'affirmer que le recul de l'âge de départ à la retraite fait partie intégrante de la concertation ... Finalement, s'agit-il d'une cacophonie ou bien d'un jeu de rôles savamment orchestré ? M. le Premier ministre a affirmé hier qu'il ne reviendrait pas sur l'âge de départ à la retraite, tout en précisant qu'il faudrait néanmoins s'interroger sur un allongement de la durée du travail, propos repris, peu ou prou, ce matin même par le Haut-Commissaire. Quelle confusion ! Ma question est simple : existe-t-il, dans votre gouvernement, une volonté clairement établie et partagée de maintenir ce droit, à nos yeux non négociable, notamment pour ceux qui sont entrés tôt dans le monde du travail et qui exercent le plus souvent des métiers pénibles ? Bien entendu, ce droit doit être assorti d'un niveau de pension suffisant

J'aimerais pouvoir répondre à votre collègue, si cela ne vous dérange pas

Le vieillissement de la population qu'il induit représente un défi majeur pour notre protection sociale et son financement, notamment pour notre système de santé et de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il nous faudra déployer des moyens financiers considérables pour la prise en charge de la dépendance, baisser le reste à charge des familles, améliorer les conditions de travail dans les Ehpad, mieux tenir compte de la prise en charge à domicile : ce sont là des objectifs que nous pouvons tous viser ensemble. Pour financer ces besoins nouveaux, nous n'augmenterons pas les impôts.

Aurait-on pu éviter les scènes de violence, les scènes de pillage provoquées par les casseurs ce samedi, lors du dix-huitième acte de mobilisation des « gilets jaunes » ? Y a-t-il eu des défaillances et un manque d'anticipation ? Faut-il appeler cela de l'amateurisme ? Toutes ces questions, les Français se les posent. Ils ne veulent plus débattre, ils ne veulent plus de discours, plus de formules médiatiques : ils veulent des actes ! Nous ne sommes plus dans le cadre d'un maintien de l'ordre classique. À la suite des événements survenus, le 1 décembre dernier, à l'Arc de Triomphe, nous attendions déjà, de votre part, des actes forts. Or vous n'avez rien fait de plus, et ne rien faire de plus, c'est laisser faire. Aujourd'hui, aucune mesure politique ne pourra apaiser durablement la situation. Ce ne sont pas vos incantations qui calmeront le pays, encore moins le recours à l'armée. recours à l'armée. Votre « en même temps » dans le domaine régalien est un véritable échec. Il faut adopter la seule politique qui vaille : celle de la fermeté à la hauteur de la violence, celle que le Sénat vous propose depuis le mois de juin dernier. Pouvez-vous me dire à combien se chiffrent les dégâts ? Qui va les payer ? Les Français, qui verront leurs cotisations d'assurance augmenter ? Êtes-vous enfin prêt à faire payer les casseurs ? Je vous le rappelle, ma question s'adressait au Premier ministre ... Il se Êtes-vous sûr qu'avec un tel discrédit le ministre de l'intérieur est encore en mesure d'assumer sa mission place Beauvau ?

Ce sont les policiers eux-mêmes qui se sont adressés à nous pour se plaindre de n'avoir pas reçu les bonnes instructions. Samedi, nous continuerons à assurer l'ordre républicain, nous continuerons à protéger la République, parce que c'est cela que nous faisons. C'est la chienlit ! Je vous demande simplement de vous interroger : que feriez-vous à notre place ?

À l'heure où les Français sont indignés de voir leur pays exsangue, d'autres victimes, oubliées de tous, subissent les dommages collatéraux de cette crise, je veux parler ici des familles des membres des forces de l'ordre, de leurs épouses, de leurs époux, de leurs enfants. Depuis le début de l'année, on dénombre vingt-quatre suicides, dont dix-neuf au sein de la police nationale, des femmes et des hommes qui s'étaient engagés pour protéger les Français. Depuis des mois, la police essaie de maintenir l'ordre dans des manifestations chaque fois plus violentes. Les familles de ses agents subissent au quotidien, les réseaux sociaux, une agressivité telle qu'elles demandent à leurs enfants de ne plus dire que leur parent est policier ou gendarme. gendarme. Dans les cours d'école, on rejoue les scènes vues sur les écrans entre forces de l'ordre et manifestants. Dès lors, comment expliquer à un enfant qu'il n'est pas honteux d'avoir un parent qui a choisi cet engagement ?

Or, depuis le remaniement ministériel, rien n'a été mis en oeuvre pour entendre leur voix. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour protéger ces familles ? Pourriez-vous honorer la promesse de notre Président et prendre le temps de recevoir et d'écouter ces femmes ?

avec les syndicats, avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec les états-majors, au cours de laquelle je n'ai pas abordé la question de la prévention du suicide. Cette question, nous la connaissons tous, elle est particulièrement forte, inhumaine,

La jeunesse a manifesté pour le climat, donnant aux générations qui la précèdent, à la nôtre en particulier, une leçon de sagesse et de clairvoyance. Au même moment, un incendie se déclarait sur le, un pavillon italien avec à son bord des milliers de tonnes de fioul de propulsion et des conteneurs de matières dangereuses. L'Europe nous accompagne, notamment avec des bâtiments de sa flotte pour intervenir de manière curative sur la pollution. En lien avec Françoise Cartron, ma question porte, bien sûr, sur les mesures prises en réaction à la pollution pour protéger nos côtes et nos eaux. Certes- c'est l'occasion de le saluer depuis la catastrophe de l', l'Union européenne a accru la sécurité maritime par des mesures et des règles de prévention. L'adoption des paquets Erika 1, 2 et 3 et l'Agence européenne sont des outils efficaces.

trois défauts de règlement, dont un concernant la « rétention du fioul à bord ». Les principaux risques liés au transport maritime sont endigués grâce à l'Europe, qui nous a protégés. Néanmoins, une partie du chemin reste à faire.

Le ministre d'État, François de Rugy, s'est rendu sur les lieux dès jeudi dernier pour assurer, heure par heure, le suivi de l'incident, pour mettre en place les opérations de secours, pour saluer le sauvetage des vingt-sept personnes qui se trouvaient à bord et pour renforcer la lutte contre l'incendie ainsi que la sécurisation de la zone.

Le dernier contrôle date du 26 octobre 2018 à Hambourg ; en France, nous effectuons 1 600 contrôles de ce type. Si l'enquête démontrait une erreur manifeste, il faudrait bien

Nous suivons également la pollution avec un système satellitaire communautaire appelé CleanSeaNet. Une mise en demeure a été adressée à l'armateur pour qu'il mette fin aux pollutions par hydrocarbures et à la pollution par les conteneurs, et nous avons lancé une enquête administrative, judiciaire et technique pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident et en appeler à sa responsabilité. En fonction de ses résultats, nous ferons les propositions nécessaires au niveau européen pour améliorer toujours plus la sécurité et les réglementations. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour le groupe Les Républicains.

Après avoir partagé la conception de ce qu'est aujourd'hui la francophonie, c'est-à-dire cette langue française « devenue le centre de toutes les nations et de tous les peuples où elle fait souche dans sa variété », le chef de l'État a fixé un cap : apprendre, échanger et créer en français. outre, il s'est projeté au-delà de nos frontières. Il a souhaité que la France puisse, à travers son aide publique au développement, « réaffirmer son engagement fort pour l'éducation

a annoncé un nouvel élan pour les lycées français et un doublement du nombre d'élèves inscrits dans le réseau scolaire d'ici à 2025 et il a demandé à nos établissements du supérieur de s'implanter hors de nos frontières et de se regrouper en campus. L'ambition est importante. Il a également fixé de nouvelles missions aux acteurs de l'audiovisuel francophone et à nombre d'institutions qui font aujourd'hui vivre la francophonie partout dans le monde. Or, à ce jour, le volontariat international n'est toujours pas mis en place les budgets alloués aux alliances françaises comme aux lycées sont en diminution ; l'audiovisuel consacré à la francophonie est en plein doute. Alors, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire, un an après ce grand discours, quelles actions le Gouvernement conduit pour traduire les nombreux engagements annoncés ?

Tout cela sera décliné au sein des institutions européennes, afin que le français soit toujours plus et mieux enseigné aux fonctionnaires internationaux. Il est en effet essentiel, pour que l'Europe soit une réalité, que le multilinguisme y existe concrètement et que l'on puisse s'y exprimer en français. S'agissant des volontaires internationaux- une idée qui avait été mise sur la table par Mme Joëlle Garriaud-Maylam -, nous en sommes au stade de l'expérimentation, mais nous entendons bien passer au stade de l'industrialisation, si je puis m'exprimer ainsi.

ont manifesté pour que soit revue à la hausse l'ambition de la France en matière d'écologie, au lendemain de la grève de la jeunesse pour le climat. Dans les deux cas, l'inaction du Gouvernement a été fustigée. Je note que cela vous a laissé sans voix et sans réaction hier, Nicolas Hulot claquait la porte en regrettant la politique des petits pas, autrement dit l'immobilisme. Les Français vous exhortent aujourd'hui à agir. Pouvez-vous nous indiquer quelle est l'ambition du Gouvernement en matière de politique en faveur du climat et de promotion d'une écologie positive plutôt que punitive ?

vous avez cité la mobilisation des jeunes et de nos concitoyens pour le climat. Vous avez bien fait, parce que ces mobilisations sont salutaires et importantes. Nous avons besoin d'une prise de conscience

Au ministère de la transition écologique, nous sommes à la tâche tous les jours, nous n'avons pas attendu ces mobilisations pour travailler. Nous sommes déterminés. Nous avançons en matière énergétique programmation pluriannuelle de l'énergie a été présentée récemment. En 2020 fermeront les deux premiers réacteurs nucléaires en France, à Fessenheim ; nous avons signé le projet de territoire. Ce n'est pas intelligent ! D'ici à 2022 fermeront les quatre centrales à charbon qui fonctionnent encore en métropole. est en cours, elle se fait avec les territoires, que nous accompagnons. Nous créons l'Office français de la biodiversité, nous mettons en place le onzième parc naturel, nous partageons mieux la ressource en eau, au travers des Assises de l'eau, nous avons présenté

le Président de la République à Gréoux-les-Bains, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. L'enjeu de la sortie du grand débat sera aussi de proposer une feuille de route complémentaire pour être au rendez-vous de la transition écologique et solidaire.

maintes fois repoussée et on peine à en voir la ligne directrice ; la trajectoire carbone est pour le moins indécise ; le développement des énergies alternatives est balbutiant ; la sortie du nucléaire est aussi peu sereine que le dossier de la fermeture des centrales à charbon ; la fiscalité verte

conséquences de la pollution de l'air. Notre facture énergétique- 40 milliards d'euros -pèse pour plus des deux tiers du déficit de notre commerce extérieur. Alors, faites confiance à vos partenaires, les collectivités territoriales, auxquelles je vous offre une belle occasion de proposer sans délai une nouvelle grande loi Pacte II, un plan d'action pour le climat et la transition écologique. Il est temps d'agir ou Jupiter risque de devenir Éole, le dieu du vent

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement. Il a été dit

Pourquoi ? Parce qu'il est étrange que le président de l'Assemblée nationale ne défende pas les pouvoirs de contrôle

qui a menti devant une commission d'enquête parlementaire. Il est en effet établi- il suffit de lire notre rapport -que la vérité a été dissimulée devant une commission d'enquête. Notre commission a publié un rapport qui n'a donné lieu à aucune critique ; aucune de nos affirmations n'a été dénoncée. Le Bureau, souverainement et en toute indépendance,

à M. le président de l'Assemblée nationale qu'il convient de respecter strictement la Constitution pour ce qui est de nos pouvoirs de contrôle. Acte vous est

Vullien. Cet amendement vise à donner la possibilité à une région, lorsqu'elle intervient en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité par substitution, de lever un versement mobilité sur le ressort territorial de la collectivité à laquelle elle s'est substituée. Ce versement mobilité

Houllegatte. La loi d'orientation des mobilités revêt un caractère crucial pour l'avenir de notre pays. Elle doit conduire à offrir aux Français un véritable service, plus plus efficace et plus accessible, une mobilité du « porte-à-porte », c'est-à-dire une meilleure intermodalité. L'enjeu est de rendre la vie plus simple : franchir la voie rapide qui sépare la gare des arrêts de bus, passer de sa voiture ou de son vélo au TER, ne pas être confronté à des titres de transport, des tarifs et des interlocuteurs multiples pour le car, le tram, le train ... En bref, il s'agit d'éviter d'imposer un parcours du combattant à l'usager. Pour cela, il faut mettre en oeuvre une meilleure organisation des services de transports. Régions, départements, métropoles et agglomérations doivent pouvoir se réunir localement pour ne former plus qu'une seule et unique autorité organisatrice des mobilités, selon les modalités et le degré d'intégration correspondant à chaque circonstance locale. Les modes de financement de ces compétences doivent être adaptés à cette coopération renouvelée. En ce sens, l'amendement prévoit la possibilité de majorer le taux du versement mobilité, afin d'assurer une meilleure organisation des transports.

Cet amendement a pour objet d'améliorer ce suivi par le partage du secret professionnel entre AOM et organismes de recouvrement, pour permettre un échange d'informations

Par ailleurs, un travail est en cours entre les acteurs du secteur sur ces aspects d'accès aux données. Mme la ministre pourra sans doute nous apporter des précisions. Concernant le second point, la modification proposée n'aura pas d'impact dès lors que le secret professionnel ne constitue pas un obstacle à la transmission, mais

des auteurs de ces amendements, la loi n'a pas pour vocation de déterminer la validité de tel ou tel argument utilisé lors des décisions prises par l'organe délibérant d'un syndicat mixte, au sein duquel siègent les collectivités et groupements qui souhaitent y participer de façon volontaire. Par ailleurs, ces amendements sont dépourvus de portée opérationnelle, car il suffirait d'invoquer un autre motif pour atteindre le même objectif. La commission demande donc le retrait de ces quatre amendements.

Aujourd'hui, l'obligation d'un taux commun est un frein important à la mise en place de tels syndicats. En effet, au sein d'un syndicat peuvent coexister des offres de services très différentes, en fonction de la réalité des territoires. Même s'il n'y a pas forcément un lien direct entre

l'article 2 prévoit la possibilité de moduler les taux de versement mobilité par EPCI membre. Cette mesure pourrait remettre en question les équilibres financiers des syndicats mixtes existants, puisque certains EPCI

Cette modulation vise à faciliter l'adhésion à un syndicat mixte des EPCI qui y sont actuellement réticents compte tenu de l'application d'un taux uniforme de versement mobilité. Dans un certain nombre de territoires, la constitution d'un syndicat mixte permettra en effet de mieux gérer les enjeux de mobilité,

La taxe sur les meublés touristiques non classés appelée plus communément « taxe Airbnb » est affectée aux communes dans lesquelles sont localisés les meublés touristiques. Ce sont donc en majorité les villes les plus touristiques, déjà très bien loties en matière d'infrastructures de transports en commun, qui bénéficient des recettes de cette taxe. Cet amendement tend à rendre l'affectation de cette taxe plus juste, avec un partage de son produit à l'échelle régionale. Ce dispositif permettra aux régions de flécher ces nouvelles recettes, pour développer et moderniser les transports du quotidien reliant les bassins d'habitat aux bassins d'emploi, mais également pour accompagner les territoires dans leur stratégie de développement économique visant à encourager l'implantation d'entreprises en périphérie des grandes villes, dans l'objectif de diminuer les parcours domicile-travail. Ce n'est qu'en répondant à ce double objectif que nous parviendrons à désengorger la circulation, à limiter le trafic automobile et à lutter vraiment contre la pollution atmosphérique, qui atteint, vous le savez, des niveaux insoutenables dans les grandes villes de France.

est à Mme la ministre. La commission a introduit un mécanisme de solidarité en faveur des autorités organisatrices

mais il semble prématuré d'apporter une réponse de ce type. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, encore à l'instant à M. Lurel, ce sujet est en cours d'examen dans le cadre de la réflexion sur la fiscalité locale. Je propose donc la suppression de cet article au bénéfice des propositions qui pourront être faites dans ce cadre.

cet article prévoit que, en cas de faible rendement du versement mobilité, une communauté de communes pourra bénéficier d'un complément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Cela favorisera la coordination et la continuité de l'organisation des déplacements sur l'ensemble du département du Rhône. On connaît tous le millefeuille territorial, et je ne voudrais pas voir apparaître un nouveau millefeuille des mobilités. Quand on parle de mobilité au sein d'un même bassin, les limites administratives n'ont plus de sens, nos concitoyens nous le disent. En disant cela, vous l'avez compris, madame la ministre, je pense plus particulièrement aux communes iséroises du Nord-Isère situées sur l'aire urbaine de l'est lyonnais, qui sont à proximité immédiate de la gare et de l'aéroport Saint-Exupéry

Par ailleurs, elles sont bien intégrées dans le projet stratégique de la plaine de Saint-Exupéry, qui est en train de monter en puissance. Aussi, madame la ministre, au moment où vous vous apprêtez à rédiger cette ordonnance, cette ordonnance, comment peut-on examiner la situation de ces communes nord-iséroises situées à proximité de la zone de Saint-Exupéry, afin qu'elles soient bien incluses, si elles le souhaitent, dans le périmètre de ce nouvel établissement ?

Avant d'entamer l'examen de l'article 4, je voudrais souligner l'excellente coopération entre les collectivités des territoires ruraux enclavés en vue d'améliorer la mobilité. Pour les Pour les lignes d'aménagement du territoire, par exemple, communautés de communes, départements et région apportent un financement, avec l'indispensable soutien de l'État. Ces collectivités ont peu de moyens, et les efforts consentis sont considérables. que la manière dont les compagnies aériennes les traitent est inacceptable. Des sous-traitances sont mises en place, sans prendre en compte leur avis, et les conventions passées ne sont pas totalement respectées, les vols pouvant s'effectuer sur des appareils beaucoup plus vétustes que prévu, moins rapides et moins confortables. Les utilisateurs, c'est-à-dire les habitants de nos territoires, ne supportent plus de tels comportements. Je suis saisie

dont le vélo. Circuler à vélo est une possibilité ouverte au plus grand nombre, dès lors que des infrastructures et des services adaptés le permettent. Le schéma régional des véloroutes est la colonne vertébrale des aménagements cyclables au niveau régional. Sa notoriété, d'une part, et son rôle d'itinéraire magistral, notamment en entrée des agglomérations, d'autre part, en font la base des schémas locaux qui supportent la mobilité du quotidien. la mobilité du quotidien. On l'a constaté, la pratique de loisir entraîne, par porosité, une pratique de mobilité quotidienne dans les territoires. Si la région intervient rarement en qualité de maître d'ouvrage des infrastructures cyclables, il est important de souligner son rôle en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité.

de s'assurer que les futurs projets de mobilité mis en oeuvre par les autorités organisatrices compétentes tiendront compte du végétal et que les infrastructures vertes seront envisagées comme des réponses essentielles aux défis de la mobilité de demain. Le Gouvernement fait de la réussite de la transition écologique l'un des objectifs de ce projet de loi. Il convient donc de garantir la place des infrastructures vertes ou verdies dans les politiques de mobilité. Elles constituent un atout pour protéger la biodiversité, améliorer le cadre de vie et la santé des habitants, mais aussi pour favoriser l'attractivité des territoires.

de m'incliner et de suivre M. le rapporteur et Mme la ministre

La commission du développement durable a amendé ce texte afin de favoriser la coopération entre autorités organisatrices, d'assurer la cohérence des services déployés et de permettre une meilleure efficacité des politiques de mobilité. Ainsi propose-t-elle que ces bassins de mobilité soient définis et délimités à l'issue d'une phase de concertation pilotée

nous souhaitons aller plus loin, en responsabilisant toutes les parties prenantes. Ainsi proposons-nous que la carte issue de cette élaboration partenariale soit validée par le vote de deux tiers au moins des partenaires associés. dans le rapport de la commission -, « les bassins de mobilité permettront de dépasser les périmètres administratifs, pour correspondre davantage aux besoins de mobilité quotidienne des habitants ». Il convient donc que les partenaires jouent pleinement leur rôle et que chaque acteur soit responsabilisé.

Un système de validation formelle risquerait de bloquer le processus, ou en tout cas de le ralentir. Par ailleurs, il est normal que, en la matière, la région prenne ses responsabilités. Il lui incombe en effet de définir les modalités concrètes de la concertation dans l'exercice de son rôle de chef de file. L'avis est donc défavorable sur ces deux amendements

la commission, qui a souhaité renforcer la coordination et la coopération entre les autorités organisatrices de la mobilité. Nous étions d'ailleurs, en la matière, tous d'accord, car un tel renforcement est fondamental pour assurer la continuité des services de transport sans rupture de prise en charge, notamment pour les mobilités du quotidien depuis les gares et les pôles multimodaux. C'est à cette fin d'assurer la cohérence de tous les services de mobilité qu'ont été réintégrés, dans cet article, les contrats opérationnels de mobilité, qui figuraient dans l'avant-projet de loi. Ces contrats s'appliqueront à l'échelle des bassins de mobilité et devront associer toutes les parties prenantes, y compris les départements, au titre de leur compétence en matière de voirie, et les syndicats mixtes SRU, lorsqu'ils existent.

que la continuité des services de mobilité soit véritablement assurée. Ainsi, nous proposons de préciser que les contrats de mobilité auront notamment pour objectif de fixer les modalités de la coordination coordination des services organisés par les différentes AOM dans le bassin de mobilité, en particulier aux différents points de connexion entre lesdites autorités, c'est-à-dire, notamment, au niveau des gares ferroviaires et routières et des pôles d'échanges multimodaux. Quel est l'avis de la commission

Quel est l'avis de la commission ? Une nouvelle fois, laissons les AOM décider des modalités de diffusion de cette évaluation triennale. Par ailleurs, le bilan annuel fera l'objet d'une présentation devant les comités des partenaires, ce qui assure déjà une diffusion régulière de l'évaluation auprès des parties prenantes. L'avis est donc défavorable.

à établir des schémas directeurs d'aménagement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont la coordination pourra être mise en oeuvre par la région.

n° 795, présenté par M. Marchand, Ce comité sera consulté avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire, de la qualité des services et de l'information. La commission a ajouté qu'il devra être consulté au moins une fois par an, ce dont je me félicite. Mais nous souhaitons aller plus loin : notre ambition est, en présentant cet amendement, d'assurer la diversité des acteurs composant ce comité et, ainsi, de favoriser le dialogue. le dialogue. Il convient d'inscrire dans la loi la possibilité pour les AOM de fixer elles-mêmes la composition du comité des partenaires. Toutefois, celui-ci devra associer des représentants des employeurs et des associations d'usagers d'habitants, car c'est là la vocation essentielle du comité des partenaires : organiser le dialogue avec les usagers, les habitants, les employeurs. Ce sont eux les premiers concernés par les services publics mis en place, puisqu'ils en sont les bénéficiaires, les demandeurs et les financeurs. Ainsi, l'objectif est d'assurer un dialogue de proximité, à l'image de ce qui existe déjà pour les conseils de quartier, pour permettre à chacun de participer à l'évolution des mobilités du quotidien. L'adoption de cet amendement permettrait également de donner aux AOM la latitude nécessaire à la mise en place d'un comité des partenaires adapté aux enjeux de leur territoire.

Pour éviter la multiplication des échelons de structures consultatives, qui complexifie la gouvernance de la mobilité sans réelle plus-value, il est proposé de supprimer le comité de desserte ferroviaire, dont le champ d'action est plus limité que celui du comité des partenaires-

organisatrices de la mobilité avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité ou de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et de l'information mise en place.

Il est chargé des politiques d'insertion, en particulier pour les demandeurs d'emploi, les personnes éloignées de l'emploi et les populations particulièrement fragiles en situation de précarité. Les départements sont particulièrement sensibles aux questions liées à l'offre de mobilité, l'insertion dans l'emploi restant pour une bonne part conditionnée aux politiques de déplacement. Enfin, force est de souligner que les départements sont également sensibilisés aux questions de politique tarifaire.

en matière d'intermodalité, soit représentée au sein de chaque syndicat mixte de type SRU existant sur son territoire. Ces syndicats assurent la coordination des services, la mise en oeuvre d'un système d'information

En outre, le principe de libre administration des collectivités territoriales implique de ne pas imposer à une collectivité qui n'en fait pas la demande d'être présente. La coordination s'effectuera dans tous les cas entre la région, les AOM et les différents syndicats, les contrats opérationnels de mobilité, que nous avons réintroduits, sans que la région soit nécessairement membre du syndicat mixte. Le contrat opérationnel associera les différents partenaires. En commission, nous avons examiné des amendements identiques. Nous avons donné la possibilité à une région de déléguer ses services à un syndicat mixte.

l'ensemble des partenaires sociaux, notamment des syndicats de salariés. Il est important que les nouvelles offres de mobilité ou la politique tarifaire ne soient pas faites en dehors de toute vision sociale des travailleurs et entreprises contribuant à ces services de mobilité, en particulier en Île-de-France. Il ne serait pas acceptable, par exemple, que le dumping social puisse servir de variable d'ajustement. La participation de partenaires sociaux à ce comité devra être confirmée par les mesures réglementaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1231-5. Il s'agit de sécuriser la participation par la loi, au même titre au même titre que celle des communes. Quel est l'avis de la commission ? Le comité des partenaires d'Île-de-France Mobilités comprend déjà des représentants des partenaires sociaux considérés comme représentatifs, selon le code des transports. Le projet de loi précise qu'il comprendra des représentants des communes ou de leurs groupements par parallélisme avec le comité des partenaires institué

Comme je l'ai déjà indiqué hier, la gouvernance déséquilibrée d'Île-de-France Mobilités est source de lourdes difficultés entre les départements en matière d'investissement dans les transports.

les embouteillages sont un gâchis -et un enjeu environnemental si nous voulons réduire la pollution. Pourtant, Paris et la petite couronne continuent à accaparer les investissements et les transports en commun. C'est déraisonnable ! Il faut donc revoir la gouvernance d'Île-de-France Mobilités, où la Ville de Paris est surreprésentée.

les administrateurs parisiens semblent avoir des difficultés à se rendre disponibles pour les réunions. Peut-être faudrait-il les soulager ... Cet amendement vise donc à faire en sorte que le nombre de sièges de la Ville de Paris et de chaque département soit établi à la proportionnelle du nombre d'habitants.

Ensuite, il faut bien voir de quoi nous parlons. Au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités, il y a cinq représentants de la Ville de Paris. D'ailleurs, ils émanent de divers groupes politiques ; ce ne sont pas des représentants de la maire de Paris.

opposants à la présidente de région, présidente de l'autorité organisatrice, au sein du conseil d'administration. Et il y a un représentant par département, en fonction des majorités de chacun. Si nous

Cet amendement s'inscrit dans la continuité du précédent. Par leur contribution au titre du versement transport, les entreprises sont les principaux financeurs d'Île-de-France Mobilités.

me semble-t-il, modifier sans concertation des équilibres aussi subtils que ceux qui existent au sein du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités. Le Gouvernement

intercommunal. Un tel schéma régional pourra faciliter l'utilisation des vélos sur de longues distances et assurer une meilleure coordination des axes

à créer un nouvel article relatif au développement des infrastructures cyclables, avec l'instauration d'un schéma régional des véloroutes, sous la responsabilité des régions. Notre rapporteur a refusé ces amendements en commission, considérant que son amendement instaurant un schéma national des véloroutes était suffisant. Il estimait alors que les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires se chargeraient d'identifier en cohérence avec le schéma national des véloroutes et voies vertes les itinéraires d'intérêt régional à à développer. Pour notre part, nous pensons que la disposition introduite par le rapporteur doit être déclinée régionalement. En effet, les itinéraires invoqués par le rapporteur ne concernent pas spécifiquement le vélo, ce qui signifie que les Sraddet ne feront que reprendre les itinéraires inscrits dans le schéma national des véloroutes et voies vertes. Or notre philosophie est plutôt inverse : partir des territoires avec des schémas régionaux des véloroutes dont la somme constituerait le schéma national. En effet, un schéma à l'échelle nationale réduira nécessairement le nombre d'itinéraires cyclables. Un zoom à l'échelle régionale est indispensable pour irriguer le territoire de suffisamment d'itinéraires cyclables. J'invite donc M. le rapporteur à compléter le schéma national qu'il a inscrit dans le texte par ces schémas régionaux. Quel

d'entre nous, vise, dans l'hypothèse d'une fermeture ou du déplacement d'une gare, à favoriser la transformation du site. Il tend à obliger les propriétaires des locaux restés vacants à répondre dans un délai de trois mois à une proposition de convention de mise à disposition adressée par l'exécutif local et dans un délai d'un mois à toute demande d'information complémentaire. Ce dispositif doit permettre de favoriser la transformation de sites restés vacants, que l'on peut assimiler à des gares « fantômes » dont l'usage se limite à l'accès aux quais, certaines d'entre elles ne disposant même plus de salle d'attente. L'objectif est, par exemple, de parvenir aux solutions mises en oeuvre en Suisse, où le gérant d'un commerce, installé dans une ancienne gare, assure également la distribution des billets de train. Quel est l'avis de la commission ?

mais, assez curieusement, dans des endroits où le foncier est le plus cher. La gare d'Orsay, par exemple, n'a pas posé de problème particulier et est devenue un très beau musée. Toutes les gares du chemin de fer de la petite ceinture dans l'Ouest parisien ont été reconverties en lieux de commerce, d'animation, en restaurants et en boutiques. Or, assez curieusement, la SNCF ne s'intéresse pas

présenter l'amendement n° 537 rectifié. Cet amendement vise à permettre aux gestionnaires d'infrastructures routières d'être consultés par les autorités compétentes et de participer à la création ou au développement de pôles d'échanges multimodaux.

pour les pôles d'échanges multimodaux. Cet amendement vise à autoriser notamment la couverture par le produit du péage de ces contributions financières, ce qui permettra aux gestionnaires d'infrastructures routières de participer à la réalisation et au financement de pôles d'échanges multimodaux, notamment par la création de parkings.

dans le but de réduire le déficit chronique de l'établissement public, qui a confirmé le désengagement du gestionnaire des infrastructures sur les lignes capillaires- voyageurs et fret, classées 7 à 9 l'exigence s'impose à l'État d'engager une réflexion pour assurer la pérennisation de ces lignes, d'identifier dans un rapport remis au Parlement les modes de financement de ces lignes et de mettre les les moyens financiers nécessaires pour en assurer la réhabilitation, en particulier avant tout transfert de la propriété de ces lignes aux régions volontaires. Cet engagement pourrait utilement être pris avant l'élaboration des prochains contrats de plan État-région à l'horizon de 2020 et l'ouverture à la concurrence.

Haut Comité du système de transport ferroviaire d'établir un schéma national des dessertes ferroviaires qui serait présenté régulièrement présenté régulièrement au Parlement. La représentation nationale doit être informée au moins une fois par mandature des évolutions de l'offre de transport ferroviaire sur l'ensemble du territoire, d'autant que l'ouverture à la concurrence du service de transport ferroviaire de voyageurs va bouleverser de nombreuses pratiques et habitudes de l'opérateur historique, des autorités organisatrices de la mobilité et des usagers pour leurs déplacements personnels comme professionnels. Au lendemain de la promulgation Au lendemain de la promulgation de la loi au printemps dernier, alors qu'elle ne sera applicable qu'en 2020, la

Quant au deuxième volet, l'élaboration d'un schéma supplémentaire relatif aux dessertes et mobilités, il me semble alourdir le travail des régions, qui planifieront librement leurs services. Nous ne saisissons pas l'intérêt de prévoir qu'un tel schéma ferait l'objet d'une présentation et d'un débat au Parlement.

Parlement des dessertes décidées par les régions. J'ai bien en tête les difficultés que vous avez mentionnées, monsieur le sénateur, notamment les évolutions de la desserte du Grand Est en effet, à des travaux dans la gare de Lyon-Part-Dieu. Les dessertes qui existent aujourd'hui devront être revues après la fin de ces travaux. J'ai également en tête les concertations qui avaient été engagées dans Les Hauts-de-France. J'ai d'ailleurs demandé à la SNCF

Je souligne l'ouverture dont a fait preuve le rapporteur, puisque notre groupe a pu faire adopter un certain nombre d'amendements particulièrement importants à nos yeux. Il s'agit, notamment, de permettre une réelle prise en compte des enjeux de développement des voies navigables pour le transport de marchandises. Vous le savez, nous prônons non pas la concurrence entre les modes de transport et à l'intérieur de ces modes, mais la complémentarité et la coopération, plus utiles pour répondre non seulement aux enjeux de mobilité, mais également aux enjeux environnementaux. À ce titre, la prise en compte par le plan de mobilité du plan Climat, comme nous le proposions, nous semble être une avancée concrète pour l'environnement et la préservation de la biodiversité. Nous sommes également satisfaits que plus de temps ait été accordé aux collectivités pour mettre à jour un document au regard des nouvelles obligations.

En effet, l'accessibilité concerne une grande partie de nos concitoyens, puisque, démographiquement, nous savons que près de 25 % de la population française aura plus de soixante-cinq ans d'ici à une dizaine d'années, selon l'Insee. Il s'agit donc d'anticiper le vieillissement démographique. Le taux de prévalence du handicap, quel que soit le type de déficience, oscille entre 10 % et 15 % de toute population, selon l'OMS. Les familles sont également en quête d'accessibilité, notamment en raison des quelque 2,5 millions de poussettes circulant chaque jour. Les pertes de marchés touristiques dues à l'inaccessibilité des infrastructures varient entre 15 % et 20 %, selon la Banque mondiale. Alors que le Président de la République souhaite que le nombre de visiteurs étrangers passe de 85 à 100 millions par an, il convient de percevoir l'accessibilité comme participant au développement économique de notre nation. Parce que le droit à la mobilité s'exerce aussi par l'accessibilité des réseaux de transports publics, il appartient de l'ancrer dans les plans de mobilité, d'autant que cela relève du pilier sociétal du développement durable. Quel La modification proposée s'insère mal dans le cadre des transports, puisqu'elle porte sur la définition générale des plans de mobilité, à l'article L. 1214-1 du code des transports, et qu'elle ne correspond pas à des objectifs ou à des enjeux pris en compte par le plan. Ceux-ci sont définis à l'article L. 1214-2, qui prévoit déjà que le plan de mobilité vise le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite. L'amendement étant pleinement satisfait par le droit en vigueur,

des plans de mobilité renforcés embrassant mieux les nouvelles problématiques de déplacement et de transport. Il est ainsi précisé que ce plan est élaboré « en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population Par souci de clarté, cet amendement vise à ce que ce plan prenne également en compte les caractéristiques particulières, notamment topographiques et géographiques, des territoires.

l'un des défis du projet de loi d'orientation des mobilités est de répondre à l'urgence climatique. Madame la ministre, vous aviez même annoncé à l'occasion du débat sur les mobilités du futur, qui a eu lieu au Sénat en janvier dernier, votre volonté d'engager la transition complète de nos mobilités vers la neutralité carbone, qui est l'un des objectifs fixés par le plan Climat 2017. La France s'est engagée dans cette trajectoire dès 2005, en concrétisant dans la loi l'engagement de diviser par quatre ou cinq les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet de loi prévoit de supprimer cette mention et de la remplacer par l'objectif de neutralité carbone à l'horizon de 2050. Nous nous réjouissons de cette volonté d'éradiquer les émissions de gaz à effet de serre et de ne pas se contenter de les réduire. Cependant, il nous apparaît nécessaire de traduire cet objectif non seulement au niveau national dans la loi, mais également dans les territoires. La traduction des objectifs nationaux en termes de mobilité au niveau local passe par les plans de mobilité. Ces plans sont les documents de planification qui organisent pour dix ans la mobilité d'un territoire. Ils sont la pierre angulaire des politiques locales en matière de mobilité. Or le lien actuel entre les plans de mobilité et les objectifs climatiques à échelle nationale est insuffisant et inopérant. C'est pourquoi il nous semble nécessaire que soit inscrit dans les plans de mobilité l'objectif de diminution des émissions de gaz. Ce faisant, nous ferions des plans de mobilité des documents de planification déclinant localement la trajectoire de décarbonation des transports dans laquelle s'est engagée la France. Quel

puisqu'il régit l'organisation de la mobilité des personnes, du transport de marchandises, ainsi que la circulation et le stationnement, dans le ressort de l'autorité organisatrice de la mobilité. est élaboré en tenant compte des besoins et de la diversité de la population et des composantes du territoire. C'est pourquoi nous considérons que l'ensemble des acteurs concernés par la mobilité doit y être associé. Par conséquent, Par conséquent, nous demandons que les départements participent, aux côtés des autres acteurs, à l'élaboration et à la préparation du plan de mobilité.

à assurer « l'accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes dont la mobilité est réduite ». Le présent amendement vise à prendre en compte, outre les « territoires moins denses ou ruraux », l'accessibilité des services

Cet amendement vise à inclure le transport scolaire dans les plans de mobilité, et ce alors que près de 4 millions d'élèves sont concernés par jour. Il tend également, en cohérence avec mon amendement n° 22 rectifié, à favoriser les expérimentations de décalage des horaires d'entrée et de sortie des établissements scolaires, afin de permettre d'enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur. La redéfinition de l'offre scolaire au sein des plans de mobilité permettrait de faire des économies en réalisant autant de circuits avec moins de véhicules, de diminuer le nombre de véhicules en circulation, ce qui réduirait d'autant les émissions polluantes, et, enfin, d'améliorer les conditions de travail des conducteurs, souvent employés à temps partiel et qui verraient leur temps de travail allongé. L'exemple de la ville de Rennes est parlant : l'étalement des horaires d'entrée et de sortie des établissements scolaires a permis de désengorger les transports en commun et de réaliser des économies en optimisant l'usage des véhicules existants. La parole

présentera plusieurs avantages pour l'ensemble des acteurs, les collectivités territoriales pouvant réaliser des économies sur le coût du transport scolaire avec moins de véhicules nécessaires pour le service. La mesure aura aussi des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation.

Cela suppose une planification de l'offre d'itinéraires cyclables locaux en adéquation avec l'outil de planification de référence que constituent les itinéraires cyclables d'intérêt régional inscrits au Sraddet et les schémas vélos départementaux.

Louis-Jean de Nicolaÿ. Des itinéraires cyclables linéaires, continus et sécurisés sont indispensables à un maillage cyclable cohérent. Le report modal de la voiture individuelle vers le vélo pour des distances allant jusqu'à 15 kilomètres, voire au-delà, sera rendu sera rendu possible grâce à ce maillage du territoire local, départemental, régional et national. Les plans de mobilité doivent assurer la meilleure cohérence territoriale possible, y compris pour la circulation à vélo du plus grand nombre. Cela suppose une planification de l'offre d'itinéraires cyclables locaux en adéquation avec l'outil de planification de référence que constituent le schéma régional cyclable et les schémas vélos départementaux. Ces derniers sont établis en cohérence avec les schémas de niveau supra-européen ou national et en lien avec les acteurs publics du territoire.

et doit être compatible avec ces règles générales. Par conséquent, les amendements sont satisfaits par la combinaison du droit en vigueur et des ajouts au projet de loi, sans qu'il soit nécessaire de préciser spécifiquement que le plan de mobilité prend en compte les itinéraires concernés. J'en demande donc le retrait. Quel est l'avis

au nom de Michel Laugier. Le plan de mobilité s'arrête à la seule structuration des voies cyclables, piétonnières, ferroviaires et navigables. Il serait intéressant que le cadre réglementaire prévoie également le recensement des espaces publics aériens

Le code des transports prévoit déjà que le plan de mobilité intègre l'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération, notamment en tenant compte des besoins en surface nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes. Il ne paraît donc pas utile d'intégrer systématiquement un volet dédié à l'intégration des espaces publics aériens, d'autant que cette notion reste relativement imprécise. Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis sera défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Les auteurs de

Selon le dernier relevé du Cérema, 61 agglomérations dépassent aujourd'hui 100 000 habitants, ce qui correspond à 95 AOM soumises à l'obligation d'élaboration d'un PDU. Or les alinéas 23 et 24 de l'article 5 du projet de loi modifient cette règle pour cibler directement les AOM dont le ressort territorial comporte plus de 100 000 habitants, en supprimant la référence à la notion d'agglomération. Ce faisant, plus d'une vingtaine d'AOM, généralement de taille moyenne, se retrouveraient à basculer dans un régime d'obligation d'élaborer un plan de mobilité, car leur ressort territorial dépasse le seuil de 100 000 habitants, alors même que leur agglomération, au sens de l'Insee, comporte bien moins de 100 000 habitants. Ces nouvelles dispositions risquent de peser fortement sur ces AOM, qui sont la plupart du temps composées de nombreuses communes rurales, où la mise en oeuvre d'un plan de mobilité n'est pas pertinente. pertinente. L'amendement tend donc à revenir aux critères actuellement en vigueur, tout en orientant les AOM non soumises à cette obligation vers l'élaboration d'un plan de mobilité rurale, davantage adapté aux spécificités des AOM

ou PCAET. C'est une obligation pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Or il n'y a pas aujourd'hui de lien juridique entre les plans de mobilité, qui sont des documents de planification

simplement à rendre compatibles ces plans de mobilité, qui sont élaborés par les AOM, avec les PCAET. Il est

prévoir l'élaboration par une AOM d'un PCAET dès lors que son ressort territorial n'est pas couvert par un tel plan, cela ne nous semble pas pertinent pour deux raisons. D'abord, cette situation va se produire fréquemment, dès lors que la compétence AOM est exercée au niveau d'un syndicat mixte.

tend à imposer que le programme d'actions prévu par le plan de mobilité comporte certaines dispositions jusqu'à présent facultatives. Il prévoit également que les entreprises situées dans des zones classées UX dans le PLU -sont particulièrement visées les zones commerciales, qui ont nécessairement des caractéristiques communes, notamment en ce qui concerne les horaires de travail -, mettent en place un plan de mobilité dès lors qu'il s'agit d'entreprises de plus de 10 salariés relevant d'une zone d'aménagement concerté regroupant plus de 200 salariés. Il s'agit de réaffirmer la place des entreprises dans la gouvernance locale des mobilités, en renforçant les plans de mobilité des employeurs pour répondre de manière efficace aux besoins de mobilité du quotidien de leurs salariés. Quel

commission ? L'exigence de compatibilité entre le SCOT et le plan de mobilité unique d'Île-de-France justifie que l'on consulte la métropole du Grand Paris, chargée d'élaborer le SCOT, sur le plan de mobilité de la région. L'avis est favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis.

Dans cette optique, l'article 5 enrichit à la fois le contenu des plans de mobilité et celui des plans de mobilité rurale créés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Afin d'améliorer la lisibilité de l'architecture des documents de planification en matière de mobilité, le présent amendement précise explicitement que les plans de mobilité rurale doivent être élaborés par les AOM qui n'ont pas l'obligation d'élaborer un plan de mobilité, à condition qu'elles n'aient pas déjà opté pour l'élaboration volontaire d'un plan de mobilité.

Nos concitoyens veulent s'exprimer, prendre part à la vie de la cité, être impliqués, ne pas subir sans comprendre. Il faut l'entendre. Le plan de mobilité sera d'autant mieux accepté qu'auront pu se croiser les avis les plus divers. La connaissance est aussi locale ; elle n'est pas seulement dans les bureaux d'études. La concertation doit être la plus large possible. Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation des parties concernées : représentants des professions, usagers des transports, associations de personnes handicapées, gestionnaires de voiries, associations agréées de protection de l'environnement, chambres consulaires, etc. Cette consultation riche permettra d'étoffer le plan de mobilité, de le rendre plus judicieux et plus efficace, ce qui est vertueux. Une telle démarche est non seulement logique, si on a le souci de l'efficacité,

de la société civile à leur demande reprend le droit en vigueur, résultant de la loi de transition énergétique de 2015. Gardons de la souplesse pour les collectivités territoriales : c'est le maître mot depuis que nous examinons ces questions. L'avis est défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Nous avons

n° 247 rectifié. L'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements exerçant certaines compétences, notamment les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité, à créer et à exploiter des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hydrides. De nombreux syndicats d'énergie de taille départementale ont ainsi entrepris de déployer des réseaux de bornes de recharge sur leur territoire. Dans le cadre de la procédure consultative, ces syndicats sont également habilités à élaborer, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, le PCAET, mentionné mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Dans le même esprit, le présent amendement a pour objet de permettre à un grand syndicat d'énergie, compte tenu de l'expérience qu'il a pu acquérir dans la mise en oeuvre de la mobilité propre et de la planification énergétique sur son territoire, d'être associé à l'élaboration d'un plan de mobilité rurale pour le compte et à la demande d'une ou de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité dont le périmètre est totalement inclus dans le sien. Il est important de préciser que le syndicat d'énergie n'a en aucun cas vocation à se substituer à l'autorité organisatrice de la mobilité, qui reste chargée d'adopter le plan de mobilité rurale, mais uniquement à lui apporter l'appui et l'expertise dont cette autorité peut avoir besoin, si bien entendu si elle le souhaite. Tel est le sens de cet amendement que je vous ai présenté au nom de mon collègue Loïc Hervé.

à l'élaboration des plans de mobilité rurale, sans préjudice des compétences des autorités organisatrices de la mobilité. Adopter cette mesure serait logique au regard du fait que ces syndicats sont déjà autorisés à élaborer le PCAET pour le compte d'un ou plusieurs EPCI.

l'initiative de Daniel Laurent et de Loïc Hervé, afin de prévoir la consultation des syndicats d'énergie actifs en matière d'infrastructures de recharge électrique sur le projet de plan de mobilité rurale. Les syndicats d'énergie sont certes des

Le transport scolaire représente une mobilité sûre et adaptée à la desserte des territoires, notamment des territoires ruraux, pour lesquels ils représentent parfois l'unique moyen de transport public.

L'ouverture de l'accès aux transports scolaires permettrait d'offrir une solution sûre et de qualité aux salariés rencontrant des difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail, et ne représenterait pas un coût supplémentaire pour la collectivité. En effet, cet amendement prévoit une compensation de la part de l'entreprise employant les salariés bénéficiaires du transport scolaire en lien avec l'autorité organisatrice de transport scolaire, selon les spécificités et contraintes de chaque territoire. Cette mesure se veut également sociale, sachant que le taux de personnes ayant déjà dû renoncer à un travail ou à une formation parce qu'elles ne pouvaient s'y rendre atteint 43 % chez les jeunes et dépasse 50 % chez les populations les plus fragiles socialement.

de l'attention que vous ne manquerez pas de porter à cet amendement dans le cadre du développement de nos territoires ruraux. Quel

vise à s'appuyer au maximum sur les transports déjà existants dans les zones rurales, en particulier le transport scolaire, qui est souvent le seul transport public régulier dans ces zones, pour développer une offre de mobilité à l'adresse des habitants de ces territoires.

Le projet de loi d'orientation des mobilités a pour objet la réussite de la transition écologique et énergétique et doit permettre de faire émerger les mobilités et infrastructures correspondantes, répondant aux besoins des populations comme des territoires, notamment en matière d'aménagement. Au-delà de ses effets directs sur la qualité de l'environnement, la végétalisation a un impact sur la physionomie de la ville et la qualité de vie : les îlots de verdure offrent au regard un paysage diversifié et procurent des espaces reposants aux habitants. Le développement des nouvelles mobilités et des infrastructures suppose de poursuivre cette logique de végétalisation des pistes cyclables, des voies de tramway et des gares ou encore de colonisation du mobilier urbain lancée par de nombreuses collectivités, telles que Le Havre, Rouen

d'après les orientations nationales, pour assurer les continuités écologiques. Par des amendements précédents, nous avons intégré la notion d'infrastructure végétale en début de projet de loi et la protection de la biodiversité dans la programmation des infrastructures. Toutefois, l'insertion de cette notion ici ne paraît pas judicieuse. Pour ces raisons,

toute dimension régénératrice de la trame verte et bleue, ce qui est incohérent avec les autres textes relatifs aux Sraddet et

parler de logistique, ce parent pauvre de la LOM : cachez cette logistique que je ne saurais voir ... Cet amendement porte sur l'implantation des plateformes logistiques, véritable enjeu d'aménagement du territoire. Ces implantations doivent reposer sur une cohérence d'ensemble, sur une planification allant à l'encontre de choix parfois trop opportunistes. Le foncier disponible ne doit pas être la seule clé de lecture. La présence d'axes de transport, leur capacité à supporter un trafic de poids lourds intense, la proximité des bassins de vie sont aussi à prendre en compte. Cet amendement vise à confier aux élus un véritable outil de planification en proposant que les Sraddet intègrent la localisation des activités logistiques, en préservant les sites existants et en prévoyant des zones futures à développer, en lien avec les besoins du territoire. Quel Quel est l'avis de la commission ? Il s'agit là encore d'un enjeu de simplification. L'article 5 du projet de loi complète déjà les objectifs de moyen et long terme du schéma en y intégrant la logistique et le développement des transports de marchandises. Or le droit en vigueur prévoit que le Sraddet comprend une carte synthétique et des règles générales en vue de mettre en oeuvre les objectifs, y compris ceux ajoutés par le projet de loi en matière de logistique et de transport de marchandises. La combinaison du droit existant et des ajouts prévus par le texte initial du projet de loi satisfait donc pleinement cet amendement, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des précisions.

Michèle Vullien, pour explication de vote.

Olivier Jacquin, pour explication de vote. pour vous interroger sur un point important. Une loi de 2013 prévoyait de doter notre pays d'une véritable stratégie logistique.

Madame la ministre, je vous ai

sont extrêmement récents. Leur nature a été clairement définie. Nous avons pris soin, en accord avec la commission du développement durable, de préciser que les plans de mobilité devaient être parfaitement articulés avec les Sraddet

présenter l'amendement n° 240 rectifié. Les usages de la voirie se multiplient et des conflits apparaissent entre des usagers qui ont des gabarits, des vitesses, des niveaux de sécurité différents. Ainsi, l'accaparement de l'espace public pour des usages privés tels que le stationnement de camions de livraison, de vélos, de trottinettes ou de voitures s'étend de jour en jour. Dans un souci de préservation de l'espace public, cet amendement tend à inciter les les porteurs de projets immobiliers à répondre, au travers de l'emprise des projets, aux besoins en livraison et expédition, afin de rendre la voirie à l'usage partagé, d'alléger la pression qu'elle subit et de limiter la congestion.

d'appel visant à attirer l'attention du législateur et des élus locaux. Dans les zones à forte pression foncière, où le prix du mètre carré est extrêmement élevé, consacrer des espaces à la logistique

Le scrutin est ouvert.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

Si les prérogatives en matière d'implantation d'espaces logistiques reviennent pour l'essentiel aux autorités communales et intercommunales, l'État peut encourager les collectivités à préserver les espaces logistiques existants et à favoriser le développement de nouveaux espaces.

et pour le schéma directeur de la région d'Île-de-France. Nous proposons de compléter le texte pour que les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intègrent la thématique du transport de marchandises, en vue de faciliter le déploiement des espaces logistiques. Quel

des activités logistiques en facilitant la transcription opérationnelle de cette planification dans les PLU. Cette transcription permettrait de préserver les sites existants, tout en prévoyant les zones à développer

plus propices. L'article 5 du projet de loi prévoit que le PLU identifie, « dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la réalisation d'équipements logistiques est nécessaire

ou rurale. Or il convient de les identifier également, dans un souci de planification et d'aménagement des territoires, les besoins des collectivités territoriales en emprises logistiques étant propres à chacune, selon ses caractéristiques. Quel est l'avis de la commission ? L'article 5 du projet de loi prévoit que le règlement d'un PLU pourra délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la réalisation d'équipements logistiques est possible. Nous ne comprenons pas clairement quelle est la distinction faite entre les secteurs dans lesquels dans lesquels la réalisation de tels équipements est nécessaire et les emprises d'activités logistiques. En tout état de cause, rien aujourd'hui n'empêche les élus d'identifier dans leur PLU des zones réservées à certaines activités économiques. Le zonage est fait pour accueillir l'ensemble des activités économiques possibles. L'avis est défavorable.

d'infrastructures cohérent. Les nombreux vols de vélo découragent largement les citoyens qui souhaiteraient trouver une alternative à l'automobile. La présence

Il s'agit de préciser dans les plans de mobilité la localisation des parcs de rabattement et des stationnements sécurisés pour vélos.

qui prévoit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou des entrées de ville, et par le projet de loi tel que modifié en commission. En effet, comme M. Jacquin y a fait allusion, nous avons décidé d'intégrer au plan de mobilité

amendement au nom de notre collègue Martine Berthet. Il a pour objet d'augmenter le nombre de trains express régionaux, mode de transport non carboné favorisant grandement la mobilité, notamment dans les zones rurales. Les citoyens doivent pouvoir se rendre sur leur lieu de travail par le biais d'une mobilité décarbonée, grâce au bon maillage territorial de notre réseau ferré et à un cadencement adéquat des trains. Alors que la SNCF a annoncé la fermeture de certaines gares et petites lignes, il est indispensable de permettre aux régions de développer l'utilisation de TER pour favoriser les déplacements des citoyens, notamment excentrés.

La portée de cet amendement n'est pas très claire. De fait, les régions prennent déjà en compte l'évolution des besoins de mobilité, sans qu'il soit nécessaire de le préciser ; c'est l'essence même de leur rôle en la matière. On ne peut pas signer une convention TER pour six ans sans s'interroger sur l'évolution des flux sur la période. Je demande

Laure Darcos, pour explication de vote.